Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l’orateur disposera alors à son tour du droit de repartie, pour une minute. Madame la ministre déléguée, vous pourrez donc, si vous le souhaitez,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la réflexion prospective est plus que jamais indispensable dans le monde où nous vivons. Il importe d’anticiper et d’imaginer différents futurs possibles, d’analyser les tendances actuelles, les facteurs de changement et de prendre en compte les incertitudes qui pourraient façonner le monde de demain. Pour cela, la planification est un outil central qui s’inscrit depuis toujours dans une tradition bien française. Déjà, en 1944, le Conseil national de la Résistance, dans ses propositions, s’inspire des politiques du plan, énonce un ensemble de principes politiques et sociaux restauration de la démocratie, égalité des droits, droit au travail, sécurité sociale, réforme du système éducatif et nationalisation de certains secteurs clés de l’économie. En 1946, le Commissariat général du plan, imaginé par Jean Monnet, s’impose comme une planification influencée par le en définissant les priorités économiques de la Nation. Il permet de reconstruire et moderniser les infrastructures, les industries et l’agriculture de la France de l’après guerre. Dès la fin des années 1970, la planification s’épuise et a moins de sens aux yeux des décideurs politiques dans une société qui se développe autour de la mondialisation, de la construction européenne, de la décentralisation, et avec l’essor des politiques libérales. C’est d’ailleurs sous le gouvernement de Dominique de Villepin que le sort du Commissariat général du plan sera scellé. À cette époque, rares sont ceux qui cherchent à s’extraire d’une mainmise du marché confortée par des politiques ultralibérales. En 2020, la politique de planification est remise au goût du jour. Sous l’impulsion du Premier ministre Jean Castex à la suite de la crise du covid 19, M. François Bayrou est nommé haut commissaire au plan et à la prospective afin d’« éclairer les choix collectifs que la Nation aura à prendre pour maintenir ou reconstruire sa souveraineté et une autonomie européenne face à l’impact des évolutions démographiques, à la grande transition écologique et aux bouleversements du numérique et de la recomposition des chaînes de valeur mondiales ». Joli programme ! Présentée comme « tout sauf un lot de consolation » par le Président de la République, cette réanimation, en fin de quinquennat, d’un commissariat au plan, par principe chargé du long terme, a laissé certains d’entre nous perplexes. Après trois ans et demi de travaux, il nous semblait intéressant de dresser un premier bilan. Je me suis plongé dans les travaux qui ont été réalisés : de nombreux sujets sont traités, mais de manière cloisonnée ; des perspectives sont tracées, mais aucune bifurcation n’est envisagée. D’un point de vue quantitatif, seize rapports ont trait à des questions d’ordre démographique, social et économique. D’un point de vue qualitatif, on retrouve des sujets certes intéressants, mais traités en silo, sans aucune transversalité ni prise en compte des défis qui nous font face. C’est d’ailleurs bien là que le bât blesse Toute prospective reste vaine si elle se limite à des réponses technosolutionnistes, si elle se maintient dans un cadre et dans la continuité de ce qui se fait déjà, sans imaginer les risques de chocs et de crises potentielles, notamment environnementales, géopolitiques, ou l’évolution des modes de vie. On le sait, notre avenir dépend des actions entreprises aujourd’hui pour préserver les ressources et les écosystèmes. Ces actions doivent être la matrice principale de nos politiques pour l’avenir. L’innovation technologique, la coopération internationale, les changements sociaux et économiques doivent s’envisager sous le prisme de la finitude de la planète. Kenneth Boulding le rappelait : « Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Aujourd’hui, il faudrait 2,7 planètes s’il était permis à chacun sur terre de disposer du niveau de vie par tête des Français. Le 2 août 2023, nous avons consommé toutes les ressources que notre planète peut régénérer en une année. Ce que l’on appelle le jour du dépassement arrivera certainement quelques jours plus tôt cette année. Tout cela, le Haut Commissariat au plan ne le prend pas en compte. Il n’a donc malheureusement pas opéré sa mise à jour, en restant bloqué sur le mode de développement des Trente Glorieuses, qui s’est construit sur la consommation de masse, alors que l’avenir est à la sobriété, à l’efficacité, à l’évolution des modes de vie, à la lutte contre les inégalités et à la justice sociale. À ce propos, la note sur le déficit du commerce extérieur est très éclairante : le Haut Commissariat effectue des plus et des moins en matière d’importations et d’exportations. Le seul angle est la balance commerciale, ne contrebalance pas avec l’impact significatif que ces productions ont sur l’environnement, que ce soit sur la perte de biodiversité, sur la pollution ou sur le changement d’affectation des sols, ici ou de l’autre côté de l’océan. 60 % de l’excédent agricole repose sur les céréales, mais, à côté de cela, la France reste extrêmement dépendante aux tourteaux de soja brésilien et aux engrais importés. Cette spécialisation de notre agriculture n’est absolument pas interrogée. Renforcer nos exportations par la course aux rendements et au moins disant n’est pas viable. Le monde agricole le paie aujourd’hui très cher. C’est pourquoi une planification écologique digne de ce nom est indispensable. Il est impératif de répondre aux enjeux d’indépendance stratégique vis à vis des pays exportateurs de technologies et d’aligner la stratégie industrielle nationale avec les objectifs climatiques et sociaux relocaliser l’emploi sur le territoire national sur toute la chaîne de valeur ; de relocaliser et contrôler les impacts environnementaux, les émissions de gaz à effet de serre des filières industrielles. Il s’agit non pas seulement de décarboner ici, mais de produire utile et durable. Un vrai changement de paradigme ! Une véritable planification doit aussi intégrer les questions d’aménagement du territoire. Je pense aux mobilités, notamment au réseau ferré, pour mieux desservir et structurer les territoires. Laisser faire le marché amène à toujours plus de concentration, et ce à tous les niveaux. Rééquilibrer notre pays demande une action publique au travers de politiques qui n’abandonnent pas des territoires et restaurent les services publics. Cette planification nécessite des investissements. À cet égard, quelle articulation y a t il entre le Haut Commissariat au plan, France Stratégie, France 2030, le secrétariat général pour l’investissement ou avec les lois de programmation budgétaire, qui ont tendance à se multiplier dernièrement ? Plutôt qu’une planification qui n’en porte que le nom, nous proposerions une véritable feuille de route associant moyen et long termes, basée sur de nouveaux indicateurs, en particulier la santé mentale et physique de nos concitoyens, c’est à dire une planification à laquelle serait associé l’ensemble de la société – citoyens, associations, syndicats et entreprises –, sur le modèle des conventions citoyennes. La planification doit être également ascendante et non pas seulement descendante si elle veut atteindre ses objectifs. Il faut se réapproprier le temps long malgré les incertitudes, construire la résilience, engager les transitions, investir dans l’adaptation tout en atténuant le réchauffement climatique. Le travail réalisé par le Haut Commissariat reste beaucoup trop imprégné par les vieux paradigmes et ne dessine pas un futur dissocié de la croissance, de l’extractivisme, de la prédation des ressources de notre planète. En bref, il ne trace pas le chemin d’un avenir durable. C’est peu dire que nous restons sur notre faim. Pour nous, la planification est essentielle pour sortir du court termisme et de ses impasses. La reconnexion aux moyen et long termes évite de toujours courir après l’actualité et d’aller de surprise en surprise, comme notre Président de

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Plan est né, à la Libération, de la volonté de refonder l’économie française sur des bases nouvelles. Il s’agissait d’accompagner l’effort de reconstruction du pays au sortir de la guerre. Le Commissariat général du plan avait pour fonction de penser l’orientation du développement économique et industriel selon les besoins, les ressources et les ambitions du pays. Dans les années 1960, cette structure est l’instrument de la modernisation technologique de l’économie française, concrétisée par le lancement de grands projets industriels : TGV, aéronautique, spatial, maillages autoroutiers, indépendance énergétique, automobile, etc. Plus récemment, après sa mise en sommeil en 2005, l’urgence écologique, l’ampleur de la désindustrialisation et la fragilité de nos chaînes d’approvisionnement dans des secteurs essentiels ont rendu nécessaire la mise en place d’une planification. C’est pourquoi un Haut Commissariat au plan et à la prospective a été remis à l’ordre du jour en 2020. Toutefois, quelques notes et quelques mois plus tard, selon la formule du journal, une question se pose avec acuité : à quoi sert ce nouveau Haut Commissariat au plan la prospective résulte t elle d’une véritable prise en compte de l’expérience de la planification depuis 1945 ? Est ce véritablement le retour de l’État stratège ? Est ce un outil au service de notre pays, dans un contexte de mondialisation, avec une France présente sur la scène internationale, sur tous les océans, forte de ses territoires ultramarins, ou plutôt un élément de communication politique ? Nous n’aurons sans doute pas la réponse ce soir. Pour notre part, il nous semble essentiel de renouer avec une véritable planification permettant de dégager des priorités de long terme claires et déconnectées des enjeux purement électoraux. Il nous semble aussi nécessaire de dégager des objectifs de moyen terme cohérents entre eux, des objectifs qui permettent d’inscrire l’action politique, administrative et législative dans le temps long. nous sommes loin ! Il nous faut aujourd’hui une véritable planification pour la transition écologique calibrée sur l’urgence climatique ; pour une politique industrielle volontariste, pas modeste et défensive ; pour une souveraineté alimentaire et énergétique ; pour le renforcement du capital humain et pour la préservation et la transmission des savoirs. Nous avons besoin d’une planification qui associe étroitement toutes les parties prenantes. La démarche de planification doit faire société. C’est une innovation qui doit être poursuivie en associant les représentants des salariés et des chefs d’entreprise, les experts, les hauts fonctionnaires, les cadres, mais aussi les associations et les élus locaux. La planification doit permettre de se réapproprier le temps long, pour que nous cessions de subir le monde en évolution. De plus, comme l’ont souligné nombre de chercheurs, les défis auxquels notre pays doit faire face sont nombreux tant la casse de nos outils de production a été profonde. Que dire encore de nos services publics, à commencer par l’école et l’université, réduits aujourd’hui comme peau de chagrin et à la merci de Parcoursup ? Si l’État souhaite orienter la politique économique et industrielle conformément aux objectifs affichés, qu’ils soient environnementaux, sanitaires ou sociaux, il ne peut se contenter de la « coopération bienveillante » des entreprises. Il ne peut oublier que les logiques et finalités des grandes entreprises privées passent avant tout par l’optimisation du profit. Or, comme cela a été souligné par François Bayrou, actuel haut commissaire au plan et à la prospective, cette institution doit servir un « projet de société » centré sur la justice sociale au travers de l’éducation et de la santé par l’aménagement des régions en vue de réduire les inégalités.

C’était vrai hier, ça l’est encore aujourd’hui. Si l’intention politique fait peu de doute, ce débat a le mérite d’appeler l’attention sur une structure passée, c’est le cas de le dire, au second plan…

Créé après la levée du premier confinement, le HCP avait pour vocation d’accompagner le plan de relance du Gouvernement afin de surmonter les effets économiques de la crise sanitaire.

puisque le premier Commissariat général du plan avait été créé en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous l’égide de Jean Monnet et Félix Gouin. Il incarnait une forme originale de planification à la française, dont les objectifs, définis en commun avec les partenaires sociaux, étaient d’orienter les investissements vers les secteurs prioritaires pour reconstruire la France. Revenant aux sources de ce qui a fait le succès du rattrapage économique de la France pendant les Trente Glorieuses, je citerai, pour mon département et ma région, l’exemple de la mission Racine,

Assainissement des zones côtières, démoustication et construction de stations balnéaires dédiées aux classes moyennes et populaires en pleine expansion : la mission Racine a permis d’équiper ce territoire alors en crise. Depuis, le contexte a radicalement changé.

Aujourd’hui, le vrai ministre du plan s’appelle Emmanuel Macron, Président de la République. Tous les grands projets stratégiques

Aucune lettre de mission ne semble avoir été donnée à cet égard au HCP. L’aménagement du territoire reste un axe essentiel pour nos territoires. Après des années de ringardisation sémantique, le mot « planification » est redevenu porteur dans le débat public.

Officiellement abandonnés en 2006, le principe de planification et le Commissariat général du plan avaient été remplacés par le Centre d’analyse stratégique, devenu en 2013 France Stratégie.

Doté d’un budget annuel de 15 millions d’euros, prélevés sur les crédits du Premier ministre, le HCP est chargé d’orienter les politiques publiques en matière de souveraineté économique, de démographie, d’environnement et de santé. « Vaste programme ! », comme aurait dit le général

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, abandonnée depuis près de vingt ans par les gouvernements successifs, l’idée de planification a été réhabilitée par le Président de la République, Emmanuel Macron, au mois de septembre 2020, 2020, la création du Haut Commissariat au plan et à la prospective, avec pour chef d’orchestre M. François Bayrou. Mes chers collègues, quatre ans après son installation, vous souhaitez, par ce débat, dresser le bilan de cette instance et évaluer son influence sur les politiques publiques. Au risque de vous décevoir, vous ne m’entendrez pas dire que ce bilan est remarquable, que son organisation doit rester inchangée ou que son influence est sans pareille. Non, vous ne m’entendrez pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Je dresserai, comme vous, je l’espère, un bilan tout en nuances de cette jeune institution. Au risque de vous persuader, mes chers collègues, je tenterai de vous convaincre que cette instance a tout son sens, si tant est qu’elle ait les moyens de ses ambitions. Avec la crise sanitaire, le dérèglement climatique et le retour de la guerre en Europe, l’idée selon laquelle nous pourrions vivre paisiblement sans nous préoccuper de l’avenir a été réduite comme peau de chagrin. À l’image de l’abondance rêvée d’une oasis dans le désert mondialisé, le mirage de la profusion s’est peu à peu dissipé, laissant ainsi s’ancrer la notion de souveraineté dans tous les domaines. Paralysés par le temps de l’urgence et soumis aux notifications instantanées de l’actualité, peut être avions nous oublié la nécessité d’anticiper, de réfléchir à long terme et de préparer l’avenir. préparer l’avenir. Cela tombe bien, c’est justement le rôle du Haut Commissariat au plan. Est ce une idée nouvelle ? Certainement pas, puisque Jean Monnet a été nommé commissaire général du plan dès le 3 janvier 1946, sous l’impulsion du général de Gaulle.

semble pas faire l’unanimité, il n’en demeure pas moins que son existence a tout son sens. J’oserai même vous dire qu’il est utile et qu’il peut l’être encore davantage. Que ce soit pour délivrer des analyses sur des sujets stratégiques ou alimenter le débat public, une telle instance de prospective est nécessaire pour notre pays. Comment la France peut elle demain assurer sa souveraineté sans disposer de données objectives ? Comment le Parlement peut il légiférer sur l’avenir sans être éclairé par des travaux indépendants et des services compétents ? Loin de moi l’idée de vouloir dénigrer le travail que nous accomplissons avec les services du Sénat, mais reconnaissons que nous n’avons pas l’apanage des rapports prospectifs. À la lecture du dernier rapport d’activité du HCP, pris séparément, certains passages peuvent laisser perplexe.

De la démographie à la géothermie, en passant par le sashimi et l’aquaculture, tout saute, tourbillonne, voltige sous nos yeux pour finir par atterrir miraculeusement dans ce rapport. Je n’ai pas le talent d’interprétation de Louis de Funès dans, mais il faut reconnaître, plus sérieusement, que le développement de l’aquaculture est un véritable sujet de souveraineté alimentaire. En 2020, chaque Français a consommé en moyenne 31,8 kilogrammes de produits d’origine aquatique et 83 % des poissons d’élevage consommés en France sont importés. Cela étant, dans quelle mesure le Haut Commissariat au plan est il influent ? Surtout, sur quels éléments peut on évaluer cette influence ? Je remarque que de nombreux points issus de son travail relatif au vieillissement de la population ont été repris dans la proposition de loi visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population. Par ailleurs, le 22 février 2023, alors qu’elle était ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier Runacher a présenté, en compagnie du haut commissaire, un plan d’action pour accélérer le déploiement de la géothermie. Il s’agit d’un sujet stratégique majeur pour notre souveraineté énergétique, sur lequel le Haut Commissariat avait préalablement travaillé, inspirant ainsi le plan d’action présenté. n’oublie pas les nombreux partenariats noués depuis 2020 avec diverses instances et la réunion des sherpas avec les principales forces sociales et économiques du pays.

! Mieux, je suis convaincu que le Haut Commissariat pourrait avoir une tout autre utilité si son organisation faisait l’objet d’une réforme en profondeur, en commençant par sa structure. Avec une équipe de dix personnes, a t il les moyens de ses ambitions ? Ne faut il pas s’inspirer davantage de l’architecture du Commissariat général du plan créé par le général de Gaulle, avec ses 160 agents ? Par ailleurs, comment mieux articuler le Haut Commissariat au plan avec les autres instances, que l’orateur précédent a énumérées et qui font de la prospective pour l’État en matière d’action publique ? Ne faudrait il pas en placer certaines sous sa houlette, afin de gagner en clarté et de mutualiser leurs moyens, ce qui serait bienvenu en cette période de recherche d’économies ? Enfin, ne serait il pas pertinent de renforcer ses liens avec la société civile en reconnaissant le Conseil économique, social et environnemental comme véritable commanditaire des travaux du Haut Commissariat au plan ?

épanoui et central dans la conduite des politiques publiques de la France.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au mois de septembre 2020, en pleine crise sanitaire, le Président de la République nommait François Bayrou au poste de haut commissaire au plan et à la prospective, à défaut de lui

pour maintenir ou reconstruire sa souveraineté et une autonomie européenne face à l’impact des évolutions démographiques, à la grande transition écologique et aux bouleversements du numérique et de la recomposition des chaînes de valeur mondiales

Nous pourrions faire un parallèle avec le secrétariat général à la planification écologique rattaché au Premier ministre : nous avons l’outil stratégique, mais pas les moyens, en d’autres termes, des présentations PowerPoint, mais pas de quoi passer à l’action Pis, la crise budgétaire est prétexte à ponctionner massivement dans les crédits de la transition écologique, lesquels sont réduits de 2,2 milliards d’euros. Revenons aux productions du maire de Pau. En trois ans et demi, le Haut Commissariat a produit une quinzaine de rapports sur différents sujets. Le rapport d’activité de cette structure est particulièrement éclairant pour mesurer la faiblesse du travail accompli. On ne comprend pas bien la plus value des documents du Haut Commissariat, comparés à ceux de France Stratégie, organe autonome également rattaché au Premier ministre, qui a succédé en 2006 au Centre d’analyse stratégique. En sus de ses fonctions, le haut commissaire est également, depuis septembre 2022, secrétaire général du Conseil national de la refondation. Cette instance de concertation peinant à déboucher sur des mesures concrètes,

l’Espagne et l’Allemagne en font une consommation plus importante rapportée à leur surface agricole utile. L’argument « quand on se compare, on se rassure » est régulièrement avancé pour ne surtout pas penser les transitions des pratiques. La culture du maïs est même encensée et encouragée, car elle permet de piéger du carbone, mais ses besoins hydriques ne sont pas évoqués. À l’inverse, le Haut Conseil pour le climat remplit son rôle en interpellant directement le Gouvernement sur ses insuffisances. Ainsi, le 2 avril dernier, il n’a eu aucune peine à dénoncer le « risque de recul de l’ambition de la politique climatique » de l’État. Au lieu de nous gargariser de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, qui tient à des effets conjoncturels comme l’inflation, nous devrions entendre cet appel et rattraper notre retard en matière de planification. À ce jour, cinq documents majeurs de planification manquent à l’appel : la loi de programmation relative à l’énergie et au climat, la stratégie française sur l’énergie et le climat, la troisième stratégie nationale bas carbone (SNBC), le troisième plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc), enfin, la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie.

que le Haut Commissariat éprouve quelques difficultés pour s’imposer comme un interlocuteur stratégique en matière d’action publique, malgré son titre honorifique, qui rappelle l’âge d’or de la planification économique après la Libération.

la France ont été présentées par le Gouvernement et le Président de la République au mois de septembre 2023 dans le cadre de la planification écologique. Nous sommes le premier pays au monde à disposer d’un plan d’action aussi précis pour respecter l’objectif de diminuer de 55 % nos émissions en 2023. Ce plan est d’ores et déjà mis en œuvre et financé pour un montant historique de 8 milliards d’euros en 2024. Pour vous répondre précisément sur les documents de planification,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme l’observe M. le haut commissaire lui même Historiquement, le Plan a toujours eu des relations difficiles avec les gouvernements. ». Alors que nous nous penchons ce soir sur le bilan du Haut Commissariat au plan et à la prospective pour évaluer ses performances depuis sa refonte en 2020,

Le Haut Commissariat au plan, institution pivot de l’après guerre, a vu son rôle se transformer au fil du temps. Son influence s’est progressivement étiolée, ce qui a conduit à sa dissolution en 2006. Il est refondé en 2020, sa mission étant censée avoir été renouvelée. Elle est désormais axée sur les défis écologiques, technologiques et sociétaux de long terme

politiques. L’influence qu’il clame avoir exercée, notamment sur le renouveau nucléaire français, contraste avec le scepticisme public sur son rôle effectif. Cette dissonance nous conduit à interroger la méthodologie de coordination et de collaboration entre le Haut Commissariat et les autres instances décisionnelles nationales.

Comme l’a souligné à plusieurs reprises M. le haut commissaire, le Haut Commissariat au plan et à la prospective serait un « outil d’influence » plutôt que de pouvoir ou de conduite de politiques publiques.

Par ailleurs, l’implication du Haut Commissariat dans le développement d’un plan national d’action pour accélérer le déploiement de la géothermie illustre sa capacité à engager des dialogues productifs, notamment avec le ministère de la transition écologique. Cette initiative spécifique met en lumière l’importance de clarifier les modalités de contribution du Haut Commissariat

mais doivent être optimisés et coordonnés efficacement. Qui fera quoi, et avec quels moyens ? La nécessité de s’organiser et de rationaliser est impérieuse, à court et moyen termes. Le rapport de M. Jean Pisani Ferry met en évidence la nécessité urgente

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pendant plus de soixante ans, le Commissariat général du plan a structuré nos politiques publiques et piloté les grands projets menés par l’État. Aujourd’hui encore, nous bénéficions de ses réalisations en matière d’infrastructures stratégiques, telles les centrales nucléaires ou les lignes de TGV. De 1946 à 2006, ce commissariat a garanti la continuité de ces projets structurants, par delà les changements et les alternances politiques. La construction de notre parc nucléaire constitue à cet égard une réalisation unique sous la VRépublique. Voulu par le général de Gaulle, pensé sous Georges Pompidou et industrialisé sous Valéry Giscard d’Estaing, poursuivi par François Mitterrand, entretenu par Jacques Chirac et défendu par Nicolas Sarkozy, il aura finalement été sabordé par François Hollande. Heureusement, les réalisations du plan Messmer ont résisté à l’accord entre les socialistes et les écologistes. Alors que l’EPR () de Flamanville est, souhaitons le, sur le point d’être mis en service, après vingt ans de travaux et douze ans de retard, où en est l’efficacité de notre planification ? Rappelons que, dans les années 1980, nous parvenions à mettre en service jusqu’à six réacteurs nucléaires par an.

qu’en renommant ainsi l’institution on a changé sa fonction. C’est à cette époque que de nombreux dirigeants politiques et économiques se sont fourvoyés en poursuivant le mirage d’une France sans usines. On pensait alors que notre pays, où l’on est forcément plus intelligent que les autres, pourrait rester un centre de décision en cessant d’être un site de production. Il aura fallu une succession de crises sans précédent pour que nous revenions à la raison et que nous retrouvions l’urgence du temps long. Avec la crise sanitaire, la crise énergétique et la guerre en Europe, notre pays redécouvre l’impérieuse nécessité de bâtir des politiques publiques par delà les cycles électoraux. Pour réindustrialiser le pays, faire émerger des innovations de rupture, relancer un programme nucléaire ambitieux, garantir notre indépendance sanitaire, mais aussi pour assurer notre souveraineté alimentaire et renforcer notre arsenal militaire, nous devons fixer des objectifs et construire des stratégies. Dans cette perspective, tout ce qui contribue à inscrire le débat politique dans le temps long, tout ce qui permet de l’extraire des querelles politiciennes, sert les intérêts de la France. est, j’en suis sûre, tout l’objet de ce débat. Je n’imagine pas que nos collègues écologistes, qui nous rappellent sans cesse – et avec raison – l’urgence du défi climatique et la nécessité de la planification écologique, aient pu céder à quelque tentation politicienne en proposant ce débat sur le Haut Commissariat au plan

Est ce à dire que l’action du Haut Commissariat au plan et à la prospective suffit pour renouer avec la France des grands projets industriels ? Certainement pas ! Il manque même l’essentiel, selon moi.

comme s’il regardait désormais la planification comme une chose très lointaine, sur laquelle on n’aurait plus prise. C’est malheureusement le cas. La comparaison avec la Chine est, à cet égard, très instructive. Les Chinois sont devenus les champions de la planification. Ils ont fait ce qu’ils savent faire : ils ont copié une idée produite chez nous, la planification, pour l’industrialiser chez eux. Dans ce pays, lorsque l’objectif est fixé, tout l’appareil d’État se mobilise d’un coup. Le génie chinois ! La planification à la française ne doit pas déterminer tous les aspects de la société,

qu’à garnir des bibliothèques, si nous n’en tirons aucune leçon en termes de politique publique, la France se condamne elle même au déclassement. Nous sommes, je l’espère, entrés dans l’âge du « faire ». Il faut désormais nous ressaisir, non pas en ressassant des rapports, mais en les mettant en application et en mettant notre appareil productif au service de cette planification. En France, on n’a pas de pétrole, vous le savez, mais on a des idées. Il faut désormais les mettre en œuvre ! La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier sincèrement le groupe écologiste d’avoir pris

également capable d’aller au delà du simple diagnostic, pour anticiper et se montrer force de proposition. C’est ce que le Haut Commissariat au plan et à la

sur l’électricité ? Cette note évoquait une augmentation importante de la consommation électrique à venir et invitait par conséquent à mettre en œuvre un nouveau mix énergétique, fondé sur un équilibre entre les énergies renouvelables au caractère intermittent, la production d’électricité pilotable et décarbonée, donc essentiellement d’origine nucléaire, et l’engagement d’économie d’énergie. Cette note était d’autant plus pertinente qu’elle alertait sur le risque de black out, risque de black out, menace devenue particulièrement concrète un an plus tard, quand la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine s’est ajoutée aux problèmes de corrosion sous contrainte d’une partie de nos réacteurs nucléaires. En matière de géothermie également, le Haut Commissariat au plan et à la prospective a eu un effet d’entraînement certain, puisque sa note sur le sujet d’octobre 2022 a été partiellement de la géothermie lancé par le Gouvernement au mois de février 2023. Sur d’autres sujets, le Haut Commissariat au plan et à la prospective peut en revanche difficilement formuler des réponses à court terme, tant les perspectives dressées s’inscrivent dans le temps long. Je pense par exemple à la note de décembre 2020 sur les produits vitaux et secteurs stratégiques, réactualisée en 2021 et en 2023. invite le Gouvernement à adopter des politiques ciblant des filières particulières, telles que l’aquaculture, pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, agricole et industrielle. Il serait injuste de reprocher au Haut Commissariat au plan et à la

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le débat qui nous réunit ce soir pourrait se résumer ainsi : quelle est au fond l’utilité du Haut Commissariat au plan Pour répondre à cette question, je prendrai l’exemple d’un enjeu crucial pour l’avenir de notre pays : l’accès aux médicaments, dans un contexte de pénurie régulière, liée au modèle économique du système de production. Vous l’avez évoqué précédemment, madame la ministre. En 2023, 37 % des Françaises et des Français déclaraient avoir été confrontés à une pénurie de médicaments. Ces pénuries sont de plus en plus fréquentes et concernent même des médicaments aussi répandus que le Doliprane, comme l’ont relevé nos collègues Sonia de La Provôté et Laurence Cohen lors des travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur

Le haut commissaire avait d’ailleurs demandé une mission d’appui de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) sur ce même sujet, ce qui paraissait évidemment opportun

il n’a été appliqué qu’à deux aires thérapeutiques, la cardiologie et l’anesthésie réanimation, à aucune autre. Le Gouvernement n’a même pas utilisé cet indice pour identifier la vulnérabilité aux pénuries des 454 médicaments définis comme essentiels. Pourtant, des actions peuvent être menées pour lutter contre les pénuries. Il est ainsi possible de relocaliser les productions de médicaments, en particulier des principes actifs pharmaceutiques, qui représentent la phase essentielle de la production et dont dépendent les autres maillons de la chaîne de production.

pas question non plus de l’agence de l’innovation et de la souveraineté sanitaire qu’il était recommandé de mettre en place. Nous parlons ici d’un enjeu majeur. Le temps est à l’action, l’action rapide, mais pour préserver notre notre avenir. La production de rapports de prospective dans lesquels rien n’est anticipé et qui, surtout, ne sont suivis d’aucune action ne sert à rien. Les pénuries de médicaments ne sont pas à prendre à la légère. Elles créent des risques

Les parents devaient broyer un comprimé destiné aux adultes, le dissoudre dans de l’eau, puis utiliser une seringue pour mesurer la quantité adaptée au poids de l’enfant. Outre le

autre exemple significatif. Selon une étude, le risque de récidive d’un cancer de la vessie était passé de 16 % à 46 % pour les patients soignés en période de pénurie d’un traitement de référence. Enfin, les pénuries ont un coût.

aurait pu être pertinent s’il avait rendu un travail précis et concret. Il ne l’a pas fait. Pour conclure, quelle est la plus value des travaux du Haut Commissariat,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à quoi le haut commissaire au plan sert il véritablement ? Nous connaissons l’attrait du Gouvernement pour les effets d’annonce. Il s’empare de concepts et de thèmes éloquents, qui, malheureusement, se révèlent n’être que des idées creuses. Il poursuit ainsi indifféremment la même politique en ponctuant son discours de références gaullistes bien senties souveraineté », « relance », « planification », « grand débat », « refondation », « combat du siècle », « réarmement » sont autant de mots à forte portée symbolique, proclamés avec verve, mais soigneusement vidés de sens. Le président Emmanuel Macron, qui souhaitait incarner un renouveau politique, excelle en réalité dans l’une des plus vieilles pratiques politiciennes, celle de la sophistique : une apparente sagesse, mais dépourvue de réalité. La création d’un Haut Commissariat au plan est symptomatique de cette stratégie de communication. Celui ci rejoint d’autres avatars, comme le Conseil national de la refondation (CNR), le grand débat national, voire le secrétariat général à la planification écologique (SGPE). Soit ces institutions ne disposent ni de leviers de décision ni de moyens pour agir, soit elles ne sont pas décisives au moment des arbitrages. Dans son avis budgétaire sur la mission « Direction de l’action du Gouvernement », la commission des lois du Sénat déplorait la nébuleuse des entités interministérielles parmi lesquelles figure le Haut Commissariat au plan, au périmètre d’action incertain. Quelle place occupe t il en effet dans l’administration gouvernementale ? Qui peut nous dire à quoi le Haut Commissariat au plan sert véritablement ? D’abord, il ne produit pas de plan à proprement Il est tout au mieux un groupe de réflexion gouvernemental. Le terme est purement symbolique : le Gouvernement se targue d’une filiation gaulliste, mais celle ci s’arrête aux mots. Il n’a jamais été question d’une quelconque planification. La lettre de mission mentionne l’objectif d’« éclairer les choix collectifs que la Nation aura à prendre pour […] reconstruire sa souveraineté ». Le Haut Commissariat produit donc quelques notes de synthèse éparses sur des sujets divers, sans aucune cohérence ni indépendance, sans transversalité ni modernité, sans avenir ni espoir. Ce Haut Commissariat est déjà suranné, à l’image de son dirigeant. Présidant un Haut Commissariat au plan, sans plan, ce dernier est le « Don Quichotte d’une planification imaginaire », comme le résumait un journaliste. Tout cela serait anecdotique si l’existence d’une telle institution fantôme n’avait pas un coût pour nos finances publiques. Ce qui reste le plus absurde en matière de gestion des finances publiques demeure la double antenne de cette institution, séparée entre Paris et Pau, et Pau, où un bureau accueille quelques conseillers, à l’heure où la demande est urgente d’une mutualisation des moyens, notamment immobiliers. L’imposture est grossière et la déception laisse place à la colère, car c’est en réalité une occasion manquée Nous avons plus que jamais besoin de planification pour répondre aux défis de la transition écologique et énergétique, mais aussi aux enjeux économiques et sociaux, que l’on ne peut plus abandonner au gré des conjonctures, des intérêts particuliers et des visées à court terme. Nous avons besoin aujourd’hui d’une vision stratégique et politique pour définir la direction voulue, ainsi que d’objectifs à long terme. Comment, sinon, concilier l’exigence climatique et écologique avec l’activité humaine ? Comment stopper l’érosion de la biodiversité ? Comment freiner le réchauffement climatique ?

Aujourd’hui, même délocalisée à Pau, cette planification est vide de sens, de moyens et de résultats. Si vous croyez à la vertu de la planification, ne perdez plus de temps et mettez y du contenu !

» Qu’en est il vraiment et que souhaitons nous ? En 1946, lorsque le Plan a été créé sur l’initiative du général de Gaulle et de Jean Monnet, l’heure était à la reconstruction et à la modernisation du pays. L’idée de planifier l’économie française était une nécessité – une « ardente obligation », précisait le Général. Le plan quinquennal qui s’est ensuivi a assigné à chaque secteur économique des objectifs chiffrés, et ce jusqu’à la fin des années 1980. À l’évidence, nous en sommes très loin aujourd’hui. Ne comparons donc pas ce qui n’est pas comparable ! Fallait il pour autant supprimer le Commissariat général du plan en 2006, pour le remplacer par le Conseil d’analyse stratégique (CAS), devenu France Stratégie ? Le président Macron lui même le souligne : « France Stratégie mène une politique d’évaluation et non de prospective stratégique. » Tout est dit La force du Plan ne résidait pas seulement dans sa loi ou ses outils de modélisation, mais dans sa démarche prospective à moyen et long termes. Poser les bonnes questions au bon moment, apporter aux décideurs publics les solutions crédibles avaient été discutées entre tous les acteurs publics et privés, était dans l’ADN du Plan. La concertation démocratique fut l’un des éléments déterminants de la méthode de Pierre Massé. Elle est toujours et plus que jamais d’actualité. Le Plan mobilise l’expertise pour alimenter la concertation. Il doit « éclairer les choix collectifs [sur] les grands enjeux [et] sensibiliser l’opinion publique à ces sujets », écrit François Bayrou dans son rapport d’activité. À quoi ressemble le Plan en 2024 ?

C’est d’ailleurs ce rôle que s’est donné François Bayrou, répondant ainsi à la mission que lui a assignée le président Macron en 2020 : répondre aux évolutions démographiques, à la transition écologique, au bouleversement du numérique et à la reconquête de l’appareil productif. Selon vous, cher collègue Salmon, les notes et documents stratégiques du Plan n’auraient eu aucune influence sur l’action gouvernementale… Prenons le seul exemple

La pertinence du rétablissement d’une réflexion stratégique sur l’avenir de notre pays, à moyen et long termes, nous a été rappelée brutalement par la crise du covid 19. Cette crise dont l’intensité a surpris le monde entier a entraîné dans notre Nation une prise de conscience douloureuse, au delà du seul domaine sanitaire. En mettant en lumière certaines faiblesses structurelles de notre pays, elle nous a conduits à réfléchir au projet de société que la France souhaitait construire et défendre, pour elle même et face au monde. C’est la mission qui a été confiée au Haut Commissariat au plan par le Président de la République : enraciner à nouveau les défis de long terme dans le débat public. Le Haut Commissariat au plan, c’est donc avant tout une certaine conception de l’action publique notre pays, en ce moment de doutes et de grandes menaces, à trouver un chemin de souveraineté et de puissance. Cette réflexion sur un temps plus long permet à cette instance autonome de s’affranchir de la dictature de l’urgence et de la tyrannie de l’immédiat, auxquelles les décideurs politiques sont trop souvent soumis. La réflexion prospective permet une respiration bienvenue face à l’apnée que semble imposer, à longueur de plateaux de télévision, l’instantanéité de l’actualité et des réseaux sociaux. déléguée chargée du renouveau démocratique, j’ai une conviction : l’un des éléments clés pour faire progresser le débat démocratique en France est précisément notre capacité collective à prendre du recul, non pas pour fuir les questions délicates ou sensibles, mais au contraire pour formuler exactement le but que l’on se propose d’atteindre et trouver la manière de rassembler la communauté nationale pour y parvenir. Ce n’est pas toujours facile, je le conçois, et encore moins pour celles et pour ceux qui sont en responsabilité. C’est la raison pour laquelle le rôle du Haut Commissariat au plan est précieux pour notre démocratie. Il éclaire les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux qui nous font face, qu’ils soient démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires ou culturels. Des épidémies à la pénurie de médicaments, de la désindustrialisation à l’avenir de l’agriculture, de la démographie à la dette et à la question des retraites, le Haut Commissariat au plan a eu à cœur depuis sa réinstallation de prendre à bras le corps des sujets aussi sensibles qu’essentiels pour notre avenir, des sujets qui nous permettent de faire Nation et de conforter la puissance de la France dans la durée. L’ensemble des rapports produits proposent des orientations stratégiques claires et opérationnelles assorties, le cas échéant, d’éléments de planification. J’en profite pour remercier le haut commissaire, M. François Bayrou, et ses équipes de l’important travail accompli ces trois dernières années. Je terminerai en soulignant l’importance de la mission de pédagogie du Haut Commissariat au plan.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, remercie toutes et tous de votre participation à ce débat qui aura au moins eu le mérite d’inciter la plupart d’entre nous à consulter la quinzaine de rapports rendus par le haut commissaire au plan en trois ans. Cela ne nous aura pas pris trop de temps ! Le haut commissaire au plan est donc « chargé d’animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l’État et d’éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels

le plan national d’adaptation au changement climatique., notre haut commissaire au plan ne devrait pas chômer pour éclairer tous ces travaux, d’autant que nous ne manquons pas d’opérateurs ou d’autorités indépendantes qui produisent de nombreux rapports très fournis : l’Insee, la Cour des comptes, le Haut Conseil pour le climat le Cese, et j’en oublie. La prospective et l’analyse ne manquent pas dans les services de l’État ! La question sous jacente que de nombreux orateurs et oratrices ont eu le loisir de soulever est donc la suivante : à quoi sert le Haut Commissariat au plan ? Madame la ministre, je suis au regret de vous le dire : vos réponses et non réponses tout au long de ce débat n’ont pas permis de répondre très concrètement à cette question. Mon collègue Daniel Salmon l’a souligné en introduction : notre pays n’a jamais eu autant besoin de planification. Si, au sortir de la guerre, c’était la reconstruction du pays qui justifiait cet effort

Quand même le Gouvernement renonce à avoir un plan, il est difficile pour le haut commissaire au plan de se sentir investi de sa mission ! Il y a moins d’un mois, nous avons débattu dans cet hémicycle du rapport de la Cour des comptes, qui, au long de ses plus

ces opérateurs sont nombreux et produisent un travail de qualité, mais ils sont souvent ignorés et mal coordonnés avec les politiques gouvernementales. Par ailleurs, une question majeure nous taraude, celle de la démocratie. Si la planification a une histoire forte de verticalité en France, la nomination du haut commissaire au plan n’y a pas échappé. Il semble que ce mode de nomination, fait du prince par excellence, peut expliquer la défiance à son égard. Si nous devons planifier notre avenir commun, il est temps d’associer la société civile, les citoyens, le monde économique, les collectivités territoriales et le Parlement dans un effort commun et partagé pour une vision de long terme. En matière de planification, tout ne saurait être décidé à Paris un tableur Excel. Nous avons besoin d’une vision partagée, à moyen et long termes, pour faire face aux enjeux qui viennent. S’il nous faut repenser la fonction de haut commissaire au plan comme grand chef d’orchestre de cette planification, la première urgence est de repenser sa légitimité démocratique. Aujourd’hui, elle est quasi nulle. Dans un idéal logique, le haut commissaire au plan, investi par le Parlement, coordonnerait réellement les différentes stratégies de planification et viendrait régulièrement